opportunité de croissance et de développement » a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

: La parole est à Mme la secrétaire d'État. Le présent amendement, qui résulte d'un travail approfondi et conjoint avec le rapporteur Jean-François Husson, que je remercie, vise à protéger les investisseurs contre les fraudes constatées en matière d'actifs numériques, au travers de l'interdiction du démarchage pour les intermédiaires en crypto-actifs qui n'auraient pas été agréés par l'AMF. à proscrire les publicités qui seraient en réalité un démarchage dissimulé. En revanche, l'interdiction totale de la publicité pour les prestataires n'ayant pas reçu d'agrément ou de visa de l'AMF ne paraît pas nécessaire. Elle risquerait en effet de représenter un obstacle important au développement du secteur, dans la mesure où il n'existe pas de modèle économique viable pour certains de ces acteurs sans la possibilité de recourir à la publicité. Cela irait donc à l'encontre de la logique d'un dispositif fondé sur l'optionalité, qui implique de ne pas interdire, à ce stade, les projets n'ayant pas obtenu de visa.

consiste évidemment à tenir le grand public à l'écart des offres non régulées, compte tenu de la multiplication des cas de fraude recensés par l'AMF. Il s'agit en même temps d'interdire le démarchage et le parrainage, tout en assouplissant l'interdiction de la publicité, pour ne viser que les procédés utilisés par les fraudeurs. On arrive ainsi, je crois, avec cet amendement du Gouvernement, à un point d'équilibre. La commission spéciale

ces PME à la croissance extrêmement forte et rapide, ne saurait en effet justifier la dilution de l'objet du dispositif et son orientation vers le financement de structures à l'assise financière déjà stabilisée. Le PEA-PME doit permettre l'essor de PME et non la consolidation financière des entreprises à très fort potentiel. Les aides et facilités doivent être fléchées vers les entreprises n'ayant pas accès au financement privé, et, en ce sens, cette mesure diluera la portée effective de ce financement des PME sans que cela paraisse justifié. Les auteurs du présent amendement considèrent qu'il est plus juste et plus efficace, sur le plan économique, de concentrer cette capacité de financement de l'économie vers des structures en ayant véritablement véritablement besoin. Les « licornes » jouent un rôle important dans le tissu économique français, et leur croissance doit être encouragée, mais le PEA-PME n'est simplement pas le bon outil pour ce faire, d'autant que cela se traduirait par la fragilisation de PME dépendant, pour leur essor, de ce financement.

aux radars. Il y a ainsi beaucoup moins d'ETI aujourd'hui en France qu'en Allemagne, et c'est l'un des facteurs de notre difficulté à réindustrialiser le pays. Les titres de toute société ayant eu une capitalisation boursière inférieure à un milliard d'euros au cours des cinq derniers exercices seront ainsi éligibles

en raison des contraintes d'investissement que le PEA-PME représente et de son univers d'investissement réduit. Pour remédier à ce problème, l'article 27 du projet de loi introduit des possibilités de dans dans le cadre du PEA-PME. Aujourd'hui, un investisseur ne peut pas financer un projet participatif en son PEA, car il est quasi impossible de loger des actifs représentatifs de dettes, tels que des bons de caisse, dans un PEA ou dans un PEA-PME. Cet article, qui ouvrira le PEA-PME aux titres participatifs en modifiant le 1° de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, mérite d'être précisé pour permettre aux coopératives et aux mutuelles d'être assimilées à des sociétés

outil remplacera un instrument de financement des PME, et sera, au demeurant, porteur de coûts fiscaux à raison des dividendes distribués. Quand on veut encourager l'esprit d'entreprise et le travail, et non le récompenser, il y a d'autres dispositifs que celui que vous souhaitez mettre en place.

C'est en effet un risque lorsqu'ils sont rattachés au foyer fiscal.

d'effectuer des retraits avant l'expiration de la huitième année, sans clôture du plan en cas d'événement exceptionnel subi par le titulaire du plan ou son conjoint.

sur le revenu. À la lecture des données fiscales disponibles, il est évident que la durée de portage imposée est un problème pour les épargnants. En 2016, quelque 120 titulaires d'un PEA ont dû clore leur plan, ce qui a mis un peu moins de 4,8 millions d'euros en situation d'être imposés à 22

si le législateur a fait le choix de bloquer le plan d'épargne en actions sur huit ans, en échange d'une défiscalisation, c'est justement pour permettre de consacrer cet argent à l'investissement. Concrètement, le blocage de ces sommes fait office de sacrifice, compensé par une défiscalisation à sa sortie.

Premièrement, cela implique une imprévisibilité. À ce titre, la crise de 2008 a bien plus marqué les esprits que ce que l'on croit généralement. Deuxièmement, les réticences sont de plus en plus grandes à laisser voguer son épargne, lorsque l'on sait que la progression d'un titre en bourse est souvent liée au dernier plan de licenciement mis en oeuvre dans l'entreprise concernée. Ainsi, l'allocation de la ressource PEA est d'abord le véhicule d'une exigence de rentabilité. Or c'est précisément cette exigence de rentabilité qui crée une bonne partie des désordres de tous ordres auxquels vous êtes aujourd'hui confrontés.

alors même que le risque pris par l'épargnant en investissant en actions est supérieur. C'est d'ailleurs pour cette raison que la commission spéciale a décidé de les assouplir, en permettant aux titulaires d'un PEA ou d'un PEA-PME d'effectuer des retraits après de cinq ans, sans que cela entraîne la clôture du plan ou le blocage de nouveaux versements. Un peu de souplesse ne nuit pas au bon fonctionnement de ce type de produits ! La commission

Même s'il n'y a pas de bons ou de mauvais versements, je sais que les entreprises ont besoin d'avoir des fonds propres. C'est un diagnostic communément partagé,

des instruments financiers éligibles au plan en l'ouvrant à de nouveaux types de placements, les obligations remboursables en actions, les ORA, et les parts de fonds professionnels d'investissement. Pour résumer, il s'agit de formes hybrides d'entrées au capital d'une entreprise, loin de l'engagement formel qui peut être passé entre les fondateurs de celle-ci. Il faut reconnaître une forme de réactivité du Gouvernement, à la suite des difficultés rencontrées par le plan d'épargne en actions destiné au financement des PME, qui n'aura jamais séduit nos concitoyens. Toutefois, cette modification ne risque-t-elle pas de signer la fin de la logique présidant à une telle forme d'investissement dans les PME ? En effet, ouvrir les instruments financiers éligibles aux parts de fonds d'investissement ou aux titres de créance émis pour acquisition par le grand public, c'est prendre le risque, de notre point de vue, de réitérer l'histoire du cheval de Troie. En effet, le gestionnaire du PEA, qui est généralement une banque ou une compagnie d'assurance, ne manquera pas d'engager ses capacités d'action pour mener une OPA sur telle ou telle PME en attente de capitaux disponibles. Ainsi, l'entreprise, indépendamment de sa taille, sera placée encore un peu plus en situation de dépendance financière à l'égard de ces nouveaux actionnaires habillés en détenteurs d'un plan d'épargne en actions. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire, l'accompagnement des entreprises par les établissements de crédit par le biais de l'endettement contrôlé fait pleinement participer les banques à l'économie réelle. Mais la formule que vous proposez ne répond aucunement à cette logique,

La commission spéciale a adopté l'ouverture du PEA-PME aux obligations remboursables en actions non cotées, dans la mesure où il s'agit d'instruments très utilisés dans l'univers du capital investissement, par exemple pour surmonter les conflits de valorisation entre entre les dirigeants historiques et les investisseurs souhaitant entrer au capital. Par le présent amendement, il est proposé de compléter la mesure anti-abus, en plafonnant également l'exonération des plus-values afférentes à la cession de ces ORA ou

L'article 27 vise notamment à rendre éligibles de plein droit au PEA-PME les parts de fonds professionnels de capital investissement, les FPCI. En l'état actuel du droit, l'éligibilité de ces actifs au PEA-PME est conditionnée au respect du quota d'investissement de 75 % en titres de PME-ETI, parmi lesquels au moins les deux tiers doivent correspondre à des fonds propres ou quasi-fonds Cette obligation permet de garantir un niveau d'investissement élevé dans des titres de PME-ETI européennes, tout en offrant aux structures concernées une souplesse dans la composition de leur actif. de préserver ce dispositif, nous proposons de supprimer la mesure prévue aux alinéas 3 et 4 de l'article 27 , qui aurait pour effet de dispenser les parts de FPCI du respect du quota d'investissement en titres de PME-ETI, au risque,

à M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement vise à coordonner les dispositions autorisant le crédit inter-entreprises avec les nouvelles règles de certification prévues dans le projet de loi.

automatiquement le champ d'application de l'article 167 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article d'ailleurs élaboré au Sénat, avec le soutien du ministre de l'économie de l'époque.

même si celles-ci sortent du champ de la certification obligatoire. Une telle mesure permet une transition plus souple, au vu des exigences de certification introduites par le présent projet de loi, sans pour autant élargir démesurément le dispositif de prêts inter-entreprises. Vous l'avez compris, mes chers

Toutefois il nous paraît préférable de prévoir la possibilité, pour ces entreprises, de recourir à l'audit volontaire et allégé pour les petites entreprises, plutôt que d'imposer un audit classique. Tel était le sens des dispositions de l'article 27 , telles qu'elles ont été adoptées par l'Assemblée nationale, et qui n'ont pas été retenues par la commission spéciale.

En effet, il s'agissait de compléter le code monétaire et financier, afin d'introduire une dérogation au monopole bancaire et de créer deux statuts spécifiques pour les conseillers et les intermédiaires en financement participatif. En échange de cette facilitation pour les établissements, l'ordonnance permettait d'assurer quelques protections aux clients des plateformes de financement, notamment en matière d'information et de prévention des risques. Enfin, pour sécuriser le tout, le texte favorisait la supervision et la protection de la superstructure qu'est l'État, en donnant compétence aux associations professionnelles agréées, ainsi qu'à plusieurs institutions publiques, pour contrôler ses activités. Quel La commission spéciale a adopté une nouvelle rédaction de cet article. Il s'agit d'un outil utile aux entreprises, qui offre d'ailleurs une meilleure visibilité à leur raison d'être et ne diminue en rien les exigences applicables au financement participatif. La commission spéciale est donc défavorable à cet amendement.

Mme Laure Darcos. Cet amendement a pour objet d'encourager le renforcement des fonds propres des entreprises, qui sont trop souvent sous-capitalisées, ce qui les rend très vulnérables lors des crises économiques ponctuelles ou successives, car elles ne disposent pas de la solidité nécessaire pour réinvestir et relancer des projets. Il s'agirait dès lors d'exonérer d'impôt sur les sociétés la part de bénéfices qui serait affectée au fonds propre au-delà de la dotation obligatoire à la réserve légale. L'incitation fiscale peut être utile pour pousser nos entreprises à renforcer leurs fonds propres. Cela dit, je m'interroge sur le coût du dispositif et les éventuels effets d'aubaine. C'est la raison pour laquelle je sollicite l'avis du Gouvernement

ailleurs, la mise en oeuvre d'une telle disposition nous paraît délicate. Ne devrait-on pas prévoir d'imposer les bénéfices mis en réserve s'ils sont ultérieurement distribués ? Comment justifier que les entreprises qui investissent sans avoir précédemment mis leurs résultats en réserve ne soient pas concernées ?

une durée de trois ans, les intermédiaires en financement participatif, ou IFP, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d'un même groupe d'entreprises pour des opérations de crédit à la consommation. En vue d'améliorer le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, nous proposons, d'une part, d'obliger les IFP à fournir aux prêteurs les informations concernant les caractéristiques des projets des emprunteurs, et, d'autre part, de permettre au ministre chargé de l'économie de mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de trois ans s'il le juge nécessaire.

L'expérimentation proposée par les auteurs de cet amendement permettrait aux intermédiaires en financement participatif volontaires d'explorer un nouveau champ, celui du prêt à la consommation entre particuliers dans le cadre de communautés constituées autour des entreprises. Cette ouverture maîtrisée permettrait notamment le développement et la mise en oeuvre de technologies innovantes et renforcerait ainsi l'activité des plateformes. À ce titre, je suis favorable au rétablissement de l'article supprimé en commission, car le cadre défini me paraît équilibré et protecteur, tant pour les prêteurs que pour les emprunteurs. il me paraît important que la loi PACTE puisse faire une place à des dispositions expérimentales, associées à une évaluation rigoureuse- c'est bien légitime -, afin que nous puissions progressivement moderniser la façon de légiférer, mais surtout de financer notre économie.

Mme Éliane Assassi. Les actions de préférence, qui sont en fait des actions à droits particuliers, ont été introduites en droit français par l'ordonnance du 24 juin 2004 en s'inspirant des législations étrangères, notamment celles des pays anglo-saxons. Elles permettent entre autres à des actionnaires minoritaires, qui ont des objectifs strictement financiers et qui ne souhaitent pas s'impliquer dans la gestion de la société, d'aménager leur droit financier prioritaire pour bénéficier d'un dividende prioritaire ou d'une d'une répartition préférentielle du prix en cas de cession de la société. De plus, dans les sociétés non cotées, les actions de préférence s'adressent tout particulièrement à ce qu'on appelle des actionnaires de passage, pour qui la prise de participation est par nature temporaire. et Jean-Dominique Senard dénonce justement ce capitalisme de locataires, qui entraîne une augmentation des taux de profit, alors que, dans le même temps, le taux d'investissement diminue. L'internationalisation, la financiarisation et le court-termisme interrogent la notion même d'entreprise, puisque la logique entrepreneuriale cède le pas à une logique purement financière. Désormais, la valeur créée par l'entreprise doit servir en premier lieu les actionnaires, c'est-à-dire la rémunération du capital, dividendes ou plus-values ; c'est ce type d'actions que le Gouvernement, donc, veut favoriser, mais qui risque

au motif que celui-ci accroîtrait la dépendance des PME et ETI envers les marchés financiers. En réalité, c'est vraiment tout le contraire : les actions de préférence sont des outils privilégiés pour accueillir des investisseurs pouvant accompagner la société, en dehors des marchés financiers.

est à M. Richard Yung. Le présent amendement a pour objet l'assouplissement du régime des actions de préférence. Au regard des risques que font courir certaines dispositions adoptées par la commission spéciale, nous proposons de maintenir la part maximale des actions de préférence sans droit de vote à la moitié du capital social des sociétés non cotées. Nous proposons également de supprimer la mesure permettant aux statuts d'une société d'autoriser le conseil d'administration ou le directoire à distribuer des dividendes réservés aux détenteurs d'actions de préférence. Enfin, nous proposons que le rachat des actions de préférence ne puisse avoir lieu que sur l'initiative conjointe de l'émetteur et du détenteur.

premièrement, du relèvement du plafond que ne doit pas dépasser la part des actions sans droit de vote dans le capital, la limitation de ce plafond à 50 % n'a plus guère de sens, dès lors que peuvent être émises des actions à droit de vote multiple. deuxièmement, de la possibilité pour les statuts de déléguer au conseil d'administration la distribution de dividendes aux détenteurs d'actions de préférence, c'est là, en quelque sorte, un dispositif renforcé d'action à dividende prioritaire. Ce dispositif respecte le droit des sociétés, puisque les statuts doivent le prévoir et que l'assemblée générale doit préalablement avoir constaté qu'il existe des sommes distribuables sous forme de dividendes. Le respect du principe d'égalité entre les actionnaires est donc bien mentionné, mais il s'applique entre actionnaires détenant la même catégorie d'actions de préférence, et non de façon absolue entre tous les actionnaires. Ce dispositif permettrait de garantir une rémunération à l'investisseur détenteur des actions de préférence. S'agissant, troisièmement, et enfin, de la possibilité de rachat des actions de préférence sur l'initiative de leur seul détenteur, c'est là un élément très important pour l'attractivité. La possibilité d'un tel rachat doit être prévue par les statuts, qui doivent en fixer les conditions et limites, par exemple en prévoyant un délai minimal de détention ou bien une clause de sauvegarde en cas de difficulté de trésorerie de l'entreprise. De plus, le rachat doit s'opérer

du tribunal de commerce en cas d'opérations de fusion ou de scission. Il s'agit d'imposer cette obligation uniquement aux sociétés anonymes et aux sociétés européennes, ainsi qu'aux sociétés par actions participant à une fusion transfrontalière réalisée dans l'Union européenne. Nous proposons ainsi de reprendre une disposition prévue par le projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français.

de recourir aux délégations de compétences et aux délégations de pouvoir en matière de fusion. Nous proposons également qu'un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social puissent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion. Pour rappel, ces deux dispositions, comme celle de l'amendement précédent, figurent dans le projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français.

ou dirigeants des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, dans la mesure où de nombreux dispositifs permettant d'encourager la participation des cadres et de pratiquer des rémunérations au mérite ou à la performance existent. La parole est à Mme

de faire un pari collectif sur l'avenir, en proposant à chacun de contribuer au succès et à la croissance de l'entreprise. C'est d'ailleurs la même logique qu'il est proposé d'étendre aux administrateurs et aux membres

En l'état actuel du droit, lorsqu'une société émettrice a procédé, dans les six mois précédant l'attribution de BSPCE, à une augmentation de capital par émission de titres, le prix d'acquisition de ces titres bons doit être au moins égal au prix des titres émis à l'occasion de l'augmentation de capital- il ne peut lui être inférieur. Nous proposons d'assouplir cette disposition en prévoyant la possibilité d'appliquer une décote au prix des titres émis dans le cadre d'une augmentation de capital réalisée six mois avant l'attribution des bons. Le montant de cette décote ne pourrait alors être supérieur à la perte de valeur économique des titres depuis l'augmentation de capital. Il s'agirait donc de ramener à la valeur des titres initiaux. La mise en oeuvre de cette mesure contribuerait à rendre plus attractif le dispositif des bons de souscription et à renforcer la compétitivité de la place financière de Paris.

malmenée à l'article 29. Il est écrit, en effet, que les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont pour objectif de contribuer à l'éducation à la citoyenneté, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale- jusque-là, tout tout va bien : il semblerait que l'on ait véritablement reconnu le champ de leurs activités. S'ensuit néanmoins une restriction de taille, qui a tout de même un petit côté méprisant- je vais vous dire pourquoi

par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation

J'ai quelque difficulté à recevoir vos arguments. Vous vous demandez si ces activités doivent participer de l'économie sociale et solidaire.

confinent les activités éligibles aux secteurs de la réparation, du recyclage d'ordures ou de l'intervention auprès des personnes en difficulté. Tout cela est parfait, mais l'économie sociale et solidaire, y compris

M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement vise à intégrer les établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale dans le champ des bénéficiaires de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale L'article 29 a pour objet l'amélioration du dispositif. Introduit par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, l'agrément ESUS identifie les entrepreneurs sociaux dont l'activité est orientée de manière dominante vers la recherche d'un impact social significatif. L'économie sociale et solidaire réunit près de 200 000 acteurs : entreprises, associations ayant une activité économique, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales de l'économie sociale et solidaire. Les établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale

comme des entreprises sociales en charge de l'accès aux comptes bancaires, aux microcrédits, aux secours, et récupèrent progressivement les personnes évincées du monde bancaire par la financiarisation croissante du modèle bancaire international.

Nous proposons une autre rédaction : « Améliorer les actions de la Caisse des dépôts et consignations en faveur du développement des territoires ». En effet, nous ne sommes pas convaincus

A-t-elle eu tort d'accompagner le logement social ? A-t-elle eu tort d'accompagner l'aménagement de nos territoires ? A-t-elle eu tort, dans mon département, d'être dans une dynamique d'économie de la logistique du dernier kilomètre, qui est très favorable à l'attractivité de Paris ?

Mais quel est le problème ? Sur quel diagnostic l'idée que la Caisse de dépôt n'est pas au rendez-vous du développement des territoires

future Banque des territoires, sera au rendez-vous, comme elle l'est depuis deux siècles, pour nous permettre encore de répondre aux besoins des populations et des territoires, notamment en termes d'infrastructures lourdes ? C'est la question.

Nous voudrions avoir l'assurance que le fonds capitalistique ainsi constitué ne sera pas cessible à des parties privées autres que les salariés.

Nous le voyons, la taille du collège augmente alors que le poids des institutions représentées diminue. Pour notre part, nous partageons l'idée que la composition du conseil de surveillance doit être revue. Mais personne, sinon votre gouvernement, ne défend l'idée selon laquelle seul le poids de l'exécutif doit être renforcé. nous, cet article foule aux pieds la raison d'être de la Caisse des dépôts et consignations et participe à certaines manoeuvres et à diverses dispositions,

Monsieur le rapporteur,

Cette nouvelle composition permet également de faire entrer des représentants du personnel de la Caisse des dépôts au sein de la commission de surveillance, ce qui n'était pas le cas, et met en place des objectifs de parité dans les nominations.

Je voulais faire le même commentaire. Les déclarations un peu emportées de nos collègues communistes reposent sur des données inexactes. Additionnez les parlementaires, qui restent dans le même nombre, trois députés et deux sénateurs, et les personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, alors qu'il y aura moins de personnalités désignées par le ministre par le ministre et qu'il n'y a plus les représentants des corps de contrôle, sur lesquels je ne porte aucune appréciation- je serais le dernier à pouvoir le faire -mais qui n'étaient pas spécialement proches du Parlement. Vous constaterez que toutes les affirmations grandiloquentes que vous avez faites sont simplement inexactes.

Par ailleurs, c'est un établissement qui gère pour le compte des Français la collecte du livret A et d'un certain nombre de livrets spécifiques,

le groupe La Poste, la Banque postale et la CNP, poursuivront leurs missions existantes, avec la volonté de trouver assez naturellement un dans le financement des collectivités locales. On rapproche les réseaux de La Banque postale, qui sont parmi les réseaux les plus fins du territoire, et la Banque des territoires, construction plutôt tournée vers l'investissement et l'accompagnement des collectivités locales, avec des dispositifs d'ingénierie.

les personnes et les PME, de même que la CNP continuera à financer les assurances des Français. La CNP, comme vous le savez, est une institution publique, mais elle est cotée et opère aussi dans le secteur privé. La parole est à M. le rapporteur.

défavorable à cet amendement, l'article 31 ayant pour vocation, que je partage, de renforcer les prérogatives de la commission de surveillance en la rapprochant des fonctions d'un réel conseil d'administration.

mais prend des décisions touchant à l'approbation des comptes, le vote du budget, la validation de la stratégie. Cela me semble être la meilleure façon de préserver le contrôle du Parlement sur cet organisme.

en amont des choix stratégiques à un contrôle en aval des décisions, la suppression de la compétence de supervision prudentielle de la commission de surveillance et la fin du contrôle de l'utilisation du fonds d'épargne. L'objectif du Gouvernement est la remise en cause du statut public de la Caisse des dépôts et consignations pour le rapprocher du statut d'un établissement de crédit privé. En confiant la surveillance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le texte rapproche la gouvernance de celle d'une banque commerciale. La nouvelle entité, avec ses 1 000 milliards d'euros de bilan, risque de passer sous le contrôle direct de la Banque centrale européenne. Comment les missions d'intérêt public de la CDC seront-elles respectées ? Comment le socle de l'épargne populaire, le livret A, sera-t-il respecté, alors que ce placement fait perdre de l'argent à des millions de nos concitoyens ? Madame la secrétaire d'État, je le dis avec solennité, vous proposez une restructuration de fond de nos institutions financières publiques, sans toucher, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à la domination des marchés financiers. Les conséquences seront extrêmement lourdes. Le ministre Bruno Le Maire a répondu à l'Assemblée nationale qu'il ne fallait pas « créer de craintes inutiles mais, sans garanties formelles de votre part, notre rôle en tant que parlementaires est de savoir douter, de vous interroger, ce que nous faisons depuis le début, et surtout d'alerter l'opinion publique.

Cette commission assure désormais le contrôle permanent de la gestion de la Caisse. Elle délibère quatre fois par an sur les sujets pour lesquels elle n'est saisie qu'une seule fois, par exemple sur les orientations stratégiques de la Caisse ou encore la situation de la trésorerie. Elle délibère également sur les opérations d'investissement et/ou de désinvestissement. L'article lui octroie de nouvelles prérogatives telles que l'adoption du budget de la Caisse ou l'approbation du programme d'émission de titres de créances.

public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles. [ ...] « La Caisse des dépôts La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. « La Caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.

défavorable à l'amendement n° 627, puisque les dispositions relatives aux comités spécialisés apportent de la souplesse de gestion pour la commission de surveillance et ne remettent aucunement en cause le comité de gestion du fonds d'épargne. C'est ce que j'ai évoqué précédemment. est par ailleurs défavorable à l'amendement n° 628, car même si l'alinéa correspond essentiellement à un toilettage des dispositions en vigueur, il apporte également des améliorations.

à remplacer renforcent les pouvoirs de la commission de surveillance. Là où elle ne donnait qu'un avis consultatif, elle prend aujourd'hui une décision, valide les comptes, le budget et la stratégie, ce qui me paraît de nature à consolider les garanties du Parlement.

628 vise à revenir sur la capacité de la commission de surveillance à adresser au directeur général des observations et des avis. Cela ne me paraît pas aller dans le sens que vous défendez, à savoir une commission de surveillance et un parlement attentifs à ce qui se passe à la Caisse des dépôts

La sacro-sainte ouverture à la concurrence censée faire baisser les coûts pour des usagers devenus des clients a toujours été éphémère, quand elle n'a pas tout simplement été un mirage. Ici, il ne s'agit pas directement de ce phénomène puisque le directeur général aura toujours une mission de service public et la commission de surveillance de la CDC continuera à donner le la. Toutefois, il ne faut pas oublier que le retrait de l'État a toujours été marqué par une dégradation des conditions de travail des personnels publics et privés des administrations et entreprises « lâchées ». De plus, le maintien du caractère public de l'institution n'a jamais suffi à garantir le respect du cadre d'emploi. Je prendrai l'exemple

mais il faut bien voir ce que l'introduction du management issu du privé a donné sur les conditions de travail et les activités de plus en plus financées sur projet. L'actuel directeur du Centre national de la recherche scientifique, le taux de contractuels précaires est monté jusqu'à plus de 50 % des effectifs de l'Institut. À l'issue de sa première année de mandat au sein du CNRS, on ne peut que constater que le nombre de contractuels a aussi augmenté dans l'établissement et que le nombre de postes ouverts a, quant à lui, diminué. Étape suivante du processus, mais nous le verrons lorsque nous aborderons l'article 41, les chercheurs vont être poussés à collaborer avec le privé dans le cadre de leur recherche publique, quitte à sabrer l'indépendance de l'administration de recherche. Et cela, vous comprendrez que nous ne puissions pas l'accepter.

régie par des règles de comptabilité publique car elle n'est ni une banque ni un organisme privé. Il ne semble pas pertinent, au vu des missions de la Caisse, d'engager un alignement sur les standards privés dont l'intérêt n'est par ailleurs pas établi clairement. Tel est l'objet du présent amendement et du suivant, l'amendement n° 131.

Je précise que la Caisse publie déjà des comptes sociaux et consolidés, à la fois semestriels et annuels, en comptabilité commerciale. S'agissant des comptes consolidés, la Caisse respecte les normes IFRS. Par conséquent, les dispositions de l'article 33 n'entraîneront pas de charges supplémentaires pour l'établissement. Quel est l'avis

Enfin, la Caisse n'est pas soumise à la supervision de la BCE, en raison de ses activités spécifiques d'intérêt général.

clairement orientée dans la continuité de l'investissement pour l'intérêt général au service des territoires, de la transition écologique et énergétique. Elle intervient ainsi dans le dispositif « territoires d'industrie

J'aimerais savoir de quoi il s'agit, alors que l'indépendance de la Cour des comptes est garantie par l'article 47-2 de la Constitution. Comment arrivez-vous à rendre compatibles ces deux notions, qui me semblent extrêmement divergentes, madame la secrétaire

Une opération de plus grande ampleur devrait d'ailleurs avoir lieu avec le transfert des titres de l'État sur La Poste à l'établissement public financier. Mais l'article 36 crée, de fait, une situation nouvelle. nouvelle. Le dividende sera calculé, notamment, sur la base des critères prudentiels fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et non plus sur le modèle économique propre de l'établissement. Comment seront, dans ce cadre, prises en considération les sommes centralisées au titre de l'épargne populaire ou celles qui sont confiées en gestion sous mandat, par exemple ? Des pertes de ressources ne sont-elles pas à craindre en raison de ce changement de paramètre d'évaluation ? ? Ces interrogations sont lourdes et s'additionnent avec celles que nous avons émises sur les articles précédents. Elles nous conduisent, une fois de plus, à demander la suppression de l'article. est défavorable. Les modalités actuelles de fixation du montant du dividende ne sont pas satisfaisantes. En effet, ce montant est établi actuellement chaque année par un échange de lettres informel

La question de l'atteinte d'un certain niveau de centralisation des dépôts de l'épargne réglementée est au coeur du débat sur le devenir de la Caisse des dépôts. En effet, la centralisation des dépôts sur les livrets défiscalisés est une question majeure dans le débat relatif à l'épargne réglementée. Dans cet ensemble, le livret A présente une particularité essentielle. Produit défiscalisé, il constitue aujourd'hui un élément important des politiques publiques, puisque la collecte de l'épargne est affectée prioritairement au financement du logement social. Mais les choses sont un peu différentes pour le livret de développement durable et solidaire, et surtout pour l'ensemble de la collecte des réseaux « non historiques », leurs exigences de centralisation étant moindres que celles de La Poste et du réseau des Caisses d'Épargne. Cette non-centralisation est d'ailleurs devenue un problème pour ces établissements, gênés par le coût de la ressource.

De fait, il s'agit là d'une question centrale. En décidant de la centralisation des dépôts collectés au titre du livret A comme du livret de développement durable, nous pouvons trouver les moyens de financer les politiques publiques les plus importantes. Nous ne devons donc pas manquer de souffle à cet égard. Nous pourrions enfin mener la politique de rénovation urbaine correspondant aux exigences de construction de logements locatifs sociaux, lutter contre l'exclusion sociale et mettre en oeuvre une réhabilitation et une requalification du parc existant. Nous pourrions trouver les moyens de donner sens à la politique de la ville, pour ne citer que quelques exemples. Une ligne prioritaire de financement de la réalisation d'infrastructures socialement utiles peut être dégagée sur les ressources de la collecte de l'épargne populaire. On peut ensuite supprimer de notre droit fiscal l'ensemble des dispositions dérogatoires du droit commun concernant le financement des PME, en ouvrant de nouvelles lignes prioritaires adossées sur la collecte des livrets de développement durable. D'ailleurs, la suppression de ces dispositions dérogatoires, que nous appelons de nos voeux, permettrait de bonifier encore l'usage de la collecte de l'épargne réglementée en tendant vers des prêts à taux nul,

effet nécessaire de préciser les modalités de fixation de ces montants. Il convient en particulier de garantir que le montant fixé par le ministre ne porte pas préjudice à la capacité d'investissement de la Caisse des dépôts, notamment dans son rôle de banque des territoires, ni à sa capacité de mise en réserve financière. Vous avez évoqué, madame la secrétaire d'État, des discussions homériques, mais rien de très formel. Cet amendement prévoit que les montants fixés par décret soient soumis à l'avis conforme, plutôt qu'à l'avis simple, de la commission de surveillance. Cela garantira la véritable recherche d'un consensus entre toutes les parties prenantes, afin que la Caisse puisse pleinement jouer son rôle d'investisseur pour les territoires. monsieur le rapporteur,

et une faible transparence, puisqu'elle s'effectue par simple échange de lettres entre le ministre et le directeur général de la Caisse. Le projet de loi vise un objectif de clarification et de transparence, tout en renforçant le rôle de la commission de surveillance dans la détermination du versement.

? Je suis défavorable à cet amendement, car l'article 37 procède selon moi à une clarification de la mission de tiers de confiance, confiée à la Caisse des dépôts depuis sa création en 1806, sans en restreindre aucunement le champ. Quel est l'avis Gouvernement ? L'avis est également défavorable. La suppression de cette disposition reviendrait à fragiliser juridiquement l'ensemble des mandats aujourd'hui exécutés par la Caisse des dépôts pour le compte de personnes publiques.

et aux organismes de logement social, le caractère mutualisé de la rémunération des réseaux, qui se situe aujourd'hui à environ 0,3 % de l'encours collecté.

pour que soit précisé très clairement le terme « logement social », afin qu'il corresponde à la définition actuelle des bénéficiaires des prêts de la Caisse des dépôts et consignations prévue à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. l'habitation. Cet amendement vise tout simplement à pérenniser l'utilisation des dépôts collectés au titre du livret A pour le financement du logement social et garantir le fait que la Caisse des dépôts et consignations conservera les moyens de continuer à bonifier les prêts pour le logement très social-